prises pour son application, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a émis un avis favorable (16 voix pour, 2 voix contre et 1 bulletin blanc) à la nomination de Mme Catherine Guillouard aux fonctions de président-directeur général de la RATP. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l'article 3. La parole

du projet de loi d'habilitation comporte, lui aussi, des reculs en matière de droit du travail pour les salariés. En effet, sauf explicitation de votre part, madame la ministre, cet article, tel

de la réduction des critères de motivation lors du licenciement, de la diminution des sanctions en cas d'irrégularités, du raccourcissement des délais de recours pour les salariés en cas de contestation et, plus largement, de l'assouplissement du droit du licenciement économique et de la modification des règles concernant les contrats à durée déterminée. Cet article permet également d'étendre le contrat de chantier, notamment dans le secteur du bâtiment, le contrat de projet. Cette extension, voire cette généralisation, ne saurait que créer une société d'intérimaires.

Le Gouvernement propose de créer un référentiel obligatoire des dommages et intérêts alloués par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en exclut les licenciements caractérisés par une faute de l'employeur particulièrement grave. Ce qui est en cause, c'est non pas le principe de la réparation du préjudice subi, mais bien le manque de visibilité des employeurs sur les conséquences financières des licenciements. En effet, 30 % des licenciements pour motif personnel font l'objet d'un recours, et, comme l'indique le rapport de la commission, les montants peuvent osciller d'un rapport de 1 à 620 autant de risques de contentieux qui dissuadent certaines entreprises de recruter. La mise en place d'un barème est un début de solution. Encore faut-il que d'autres promesses n'en annulent pas les effets. À cet égard, je souhaiterais avoir votre avis, madame la ministre, des organisations patronales ont manifesté leur réprobation à la suite de votre annonce d'augmenter les indemnités légales de licenciement. Votre décision prend-elle en compte l'existence de tous les autres types d'indemnités, de préavis, de congés payés, supralégales ? Je comprends que la recherche d'un apaisement avec les organisations syndicales puisse justifier cette annonce. Mais avez-vous prévu une piste de simplification ? Quoi qu'il en soit, il faut aller plus loin en matière de procédure devant les prud'hommes, en revoyant notamment les délais d'instruction, comme le proposait ma collègue Françoise Gatel dans un amendement.

écarté les gêneurs, c'est-à-dire les représentantes et représentants du personnel et les délégués syndicaux, et remplacé le juge judiciaire par un décret. Apprécier la situation particulière d'un salarié et évaluer son préjudice par décret en lieu et place d'un juge est une approche profondément choquante de la justice que je refuse de partager, et je vous invite, mes chers collègues, à faire Profondément choquante et inacceptable aussi est la possibilité, pour apprécier la cause économique d'un licenciement, de dissocier l'entreprise ou le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise. Nous avons trop d'exemples, dans nos territoires, d'entreprises appartenant à des groupes florissants, bénéficiant d'ailleurs souvent d'aides publiques, actives sur des créneaux porteurs, qui distribuent les dividendes et organisent la faillite ou la casse de leur outil au détriment de l'emploi, des salariés et du développement industriel.

J'ai également demandé au préfet d'organiser le plus rapidement possible une table ronde pour réunir tous les protagonistes. Mais sans doute les plus jeunes des salariés licenciés pourront-ils être réembauchés plus tard en CDD ou en contrats de mission renouvelables à l'envi, puisque vous comptez étendre les possibilités de CDD.

à douze mois maximum, étrangement adapté à la durée de leur futur contrat de travail. Comment, mes chers collègues, pouvez-vous adopter de telles mesures et ensuite aller à leur rencontre en les assurant que la jeunesse est votre priorité ?

Ainsi, votre collègue abandonne la mission qui doit être la sienne, celle de former au mieux les jeunes de notre pays afin qu'ils aient accès à l'emploi dans les meilleures conditions, pour littéralement les « projeter » dans plus de précarité. En élargissant grandement le recours aux contrats de mission, la précarité concernera autant les jeunes qualifiés qui seront remerciés à l'issue de leur contrat que les jeunes non qualifiés promis aux petits boulots. Comment inciter les jeunes à faire des études si la seule perspective que vous leur offrez est la précarité ? Comment réduire le chômage qui frappe- faut-il le rappeler ici ?-un quart des jeunes si la seule perspective que vous leur offrez est la flexibilité ? La flexibilité fragilise encore davantage les personnes aux avant-postes de la précarité, à savoir les jeunes, les femmes et les immigrés. En fait, il s'agit de l'extension, à tous les niveaux et dans tous les secteurs, d'un CDI intermittent. Que l'on ne s'y trompe pas porte bien le nom de CDI pour rassurer- dormez, braves gens, on s'occupe de vous ! -, mais il a le goût du CDD, favorisant l'explosion de la précarité. Comment un jeune qui entre de plus en plus tard sur le marché de l'emploi peut-il accéder à un logement, fonder une famille, avec vos contrats de mission ? C'est parfaitement impossible, vous le savez. Vous le comprendrez aisément, mes chers collègues, nous nous opposons à l'article 3.

et la rend plus complexe tant au moment de la saisine qu'au niveau de l'appel. Depuis le 1 août 2016, tout salarié doit ainsi saisir les prud'hommes au moyen d'une requête écrite, compliquée, alors que cette saisine pouvait jusqu'alors se faire oralement en se rendant au siège du conseil des prud'hommes. Cette difficulté semble dissuader le nombre de salariés de faire valoir leurs droits. Un peu partout en France, les conseils de prud'hommes le constatent. Au conseil de prud'hommes de Paris, durant la période allant d'août à décembre 2016, a été constatée une baisse de 40 % du nombre de saisines par rapport à la même période en 2015. Une forte baisse est aussi constatée du côté des prud'hommes de Bobigny, une diminution telle que la juridiction a été obligée d'annuler un bureau de conciliation sur le collège de l'encadrement par manque de demandes. Du côté des prud'hommes de Lyon- on pourrait citer de nombreux autres exemples -, on a enregistré une baisse d'environ 40 % des saisines sur la période allant du mois d'août au mois de février entre 2015-2016 et 2016-2017.

Plutôt que de vouloir à tout prix limiter les contentieux, le Gouvernement serait mieux inspiré de faciliter la reconnaissance des droits des salariés victimes de la non-application du code de travail. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, sur l'article. L'article Lamure, sur l'article. L'article 3 a pour objet de sécuriser la relation de travail, ce dont nous pouvons nous réjouir. Nous devons tout faire, en effet, pour lutter contre la dualité du marché du travail qui oppose les heureux détenteurs d'un CDI à ceux qui sont embauchés en CDD ou en contrats de travail temporaire, contrats pourtant plus coûteux pour l'entreprise, mais moins risqués en matière de contentieux. Dans une tribune publiée en mars 2016, plusieurs économistes, dont le prix Nobel Jean Tirole, avaient montré que les jeunes et les moins qualifiés étaient les « grands perdants d'un marché du travail qui exclut les plus fragiles ou les relègue dans les emplois précaires, tant les entreprises craignent d'embaucher en CDI ». Aussi, toute réforme qui contribue à faire tomber les barrières à l'embauche en CDI la bienvenue. Je regrette pourtant que le projet de loi n'ait pas prévu de pousser la logique jusqu'au bout. Prenons le cas des contrats de chantier : l'étude d'impact du projet de loi précise qu'« un tel contrat peut concerner toute opération dont dont l'objet est précisément défini, le début et la fin clairement identifiés mais dont la durée et le terme sont incertains ». Il est indiqué ensuite que « ce type de contrat ne serait pas généralisé, mais bien limité aux branches ayant conclu un accord pour la mettre en oeuvre Il est dommage d'en limiter d'office l'usage, car les chefs d'entreprise sont aujourd'hui confrontés en permanence à la gestion de projets de nature très variée, dont les contraintes sont les mêmes que celles des chantiers. Le refus de la généralisation de ce type de contrat est un déni de la réalité à laquelle sont confrontées les entreprises françaises. Au printemps 2016, la délégation sénatoriale aux entreprises avait réalisé un sondage auprès de son réseau d'entrepreneurs pour savoir quelles réformes ils jugeaient prioritaires arrivait en tête de leurs besoins l'instauration d'un CDI prédéfinissant les conditions et causes de rupture, telles que la fin d'un projet ou la fin de fabrication d'un produit. Nous devons tout mettre en oeuvre pour favoriser la souplesse du contrat de travail. Ainsi, nous favoriserons l'emploi.

dans la dynamique d'inclusion, celles-ci ont droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouvert. Mais si, au cours des dernières années, à la suite du renforcement de l'obligation d'emploi des personnes handicapées par la loi de 2005, le nombre de personnes identifiées en emploi a progressé, dans le secteur tant privé que public, elles restent cependant insuffisamment présentes en milieu ordinaire de travail, au regard de l'exclusion massive dont elles font l'objet. Elles sont davantage exposées au chômage, dont le taux atteint un niveau inacceptable avec près de 500 000 demandeurs en situation de handicap, qui le sont souvent dans des conditions très défavorables notamment en termes de durée, ce qui rend leur accès ou leur retour à l'emploi difficile. Elles sont dès lors davantage exposées à la précarité, aux minima sociaux, aux ruptures de droits et aux difficultés périphériques. Elles sont vulnérables dans l'emploi et courent un risque important de perte d'emploi, notamment dans un marché du travail très concurrentiel. Le maintien dans l'emploi n'est pas encore un réflexe dans l'entreprise, et la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement par les employeurs largement améliorable. Plus de 90 % des avis d'inaptitude sont souvent suivis d'un licenciement. Le droit fondamental à exercer un travail reste un droit fragile et insuffisamment soutenu, en dépit des dispositifs et des moyens déployés. Leur trajectoire vers et dans l'emploi reste insuffisamment sécurisée pour garantir un véritable droit au travail des personnes en situation de handicap. J'attire également l'attention sur les difficultés spécifiques d'accès, de maintien ou de retour en emploi rencontrées par les proches aidants de personnes en situation de handicap. Ces inquiétudes pour l'emploi des personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants seraient surmontées par une garantie d'accès au droit de façon à permettre le déploiement de trajectoires vers et dans l'emploi pour tous, dès l'âge de seize ans et jusqu'à l'âge de la retraite, le pilotage des politiques publiques pour l'emploi des personnes en situation de handicap, qui doit inclure les moyens de mise en oeuvre, de suivi et d'évaluation, et, enfin, une attention permanente à la meilleure manière de reconnaître les aptitudes et les compétences des travailleurs handicapés, leur capacité contributive à la vie économique. Puisque l'article 3 vise à renforcer la prévisibilité et à sécuriser la relation de travail, mais aussi à clarifier les obligations de l'employeur en matière de reclassement pour inaptitude, je proposerai des amendements visant à préciser les droits des personnes handicapées en milieu de travail ordinaire et la préservation de leur accès. La parole est à Mme Gisèle Jourda, sur l'article. Madame

un salarié peut-il s'épanouir et contribuer à la vie de l'entreprise au sein de l'inquiétant dispositif que vous proposez dans votre texte,

toutes à conforter les droits de l'employeur et à fragiliser ceux de l'employé. Je ne pense pas que cela renforce le dialogue social et sécurise les travailleurs au sein de l'entreprise. À mon sens, cela ne peut que durcir le dialogue Mon intervention porte plus particulièrement sur le dispositif prévu à l'alinéa 22, c'est-à-dire la promotion, voire la banalisation, des formes de travail précaire et atypique. Je m'explique : le travail de nuit était, jusqu'à aujourd'hui, considéré par la loi et la jurisprudence comme « ayant un caractère exceptionnel Il n'est pas un mode normal d'organisation du travail et ne doit, à ce titre, être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable au fonctionnement de l'entreprise. Je pensais cette affirmation partagée par le plus grand nombre d'entre nous dans cet hémicycle. Il semble bien que non. Je me rends tristement compte que cette conception du travail, cette conception de l'exceptionnel, est celle-là même qui nous divise. Avant, nous aurions été nombreux à dire qu'il était indispensable, pour préserver la santé et la sécurité des salariés, de maintenir le caractère exceptionnel du travail de nuit. Car son caractère gravement nuisible à la santé est avéré depuis longtemps : il engendre des effets délétères sur la santé mentale et la vie sociale des employés.

Vous essayez de promouvoir un modèle que je trouve particulièrement déshumanisant pour notre société : celui de l'ubérisation, des « mini-jobs », des contrats de chantier, celui du licenciement expéditif, bref celui de la précarité. Comme si la précarité était le modèle efficace qui allait nous permettre d'affronter les mutations des trente prochaines années ... Intégrant l'infamante notion de travail effectif,

du contrat de projet ou encore le reclassement pour inaptitude. S'agissant du plafonnement des dommages et intérêts dans le cadre de licenciements sans cause réelle et sérieuse, il n'est ici question que de permettre aux entreprises de budgétiser des licenciements illégaux. Le Gouvernement opte pour la ligne dure des syndicats patronaux plutôt que pour celle des syndicats de salariés. Très bien ! Vous invoquez, madame la ministre, trois arguments. Sur 150 000 contentieux portés devant les prud'hommes chaque année, l'entreprise est paralysée par les condamnations pour vice de forme du licenciement, par les délais de jugement et par la variation du montant des dommages et intérêts pour une même ancienneté. Je suis de votre avis s'agissant du vice de forme. S'il doit être procédé aux licenciements selon les formes prévues par les lois et règlements, un vice de forme affectant une lettre de licenciement ne doit pas être automatiquement de nature entacher d'illégalité la décision prise s'il n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Je suis en désaccord, en revanche, avec la suite de votre analyse. D'abord, la durée du jugement n'est pas en lien avec l'existence ou non d'un plafond du montant de dommages et intérêts. Il est question de procédure, de stratégie contentieuse, de difficulté à rassembler les pièces, de report d'audiences, et principalement du manque de moyens alloués à la justice. Vous vous interrogez, ensuite, sur la raison pour laquelle, devant un même conseil de prud'hommes, un collègue qui était dans la même situation d'ancienneté perçoit quatre fois plus d'indemnités. La réponse est simple. La réalité d'un préjudice ne s'estime pas en fonction de l'ancienneté d'un salarié. Le préjudice peut être lié à l'âge de la personne, la difficulté à retrouver un emploi, sa qualification ou son défaut de qualification, son patrimoine, son environnement familial une cadre, veuve avec quatre enfants à charge et dix ans d'ancienneté percevra davantage de dommages et intérêts qu'une cadre avec la même ancienneté, sans enfant et mariée à un riche propriétaire. Alors, oui, il y a des écarts, et il revient au juge d'apprécier au cas par cas le montant de la réparation d'un préjudice. Je m'exprimerai sur les autres points

en vérité d'une thèse d'une grande banalité, qui a prouvé depuis longtemps son échec, mais qui est répétée. Comme le disait le juriste spécialiste de droit social Antoine Lyon-Caen, « ce projet s'inscrit dans une filiation intellectuelle [ ...] d'une grande banalité intellectuelle ».

que ces ordonnances sont une nécessité, sans apporter aucune preuve que cette logique combattra le chômage. On dit que le pouvoir se gagne par les idées c'est souvent vrai, et il est clair que, au-delà des dispositions précises de ce texte, vous menez avec ces ordonnances une bataille culturelle pour justifier la réduction des droits des salariés au nom de la prétendue compétitivité des entreprises. Ainsi, dans le texte, singulièrement dans cet article, tout est à l'avenant. Selon vous, pour rassurer les employeurs, il faudrait plafonner les indemnités prud'homales ; là encore, il faudra nous expliquer en quoi cela facilitera la création d'emplois, bien que M. Cadic, on a pu l'entendre encore à l'instant, en semble convaincu.

ce n'est qu'un CDD déguisé -, vise à nous faire prendre la souplesse attendue pour une promesse d'emplois, lesquels ne viendront jamais.

n'a jamais prouvé son efficacité pour créer des emplois. Il appauvrit les plus pauvres et enrichit les plus riches.

de travailleurs précaires, qui ont du mal à accéder au crédit, et des salariés, qui sont souvent sous le seuil de pauvreté. Comme en Allemagne, depuis les réformes Hartz,

ces ordonnances ! Les masques tombent : on donne satisfaction aux demandes les plus réactionnaires du grand patronat ! Je le dis franchement, une partie du patronat ne partage pas cette volonté de traiter ainsi le capital humain.

depuis le début de l'examen de ce texte ne nous convainquent guère, vous l'avez remarqué, et nous sommes toujours très inquiets des dangers que présente ce projet d'habilitation. Nous continuons d'essayer de faire preuve de pédagogie

plafonnement des indemnités prud'homales, la réduction du délai de recours en cas de rupture du contrat de travail, la généralisation des contrats de projets ou encore l'extension du travail de nuit, pour ne citer que quelques alinéas. Madame la ministre, pouvez-vous m'expliquer en quoi ces dispositions, qui constituent assez clairement et objectivement des reculs pour les salariés, permettent une sécurisation des relations de travail ? À moins que la sécurisation ne s'entende qu'en faveur des employeurs, auquel cas il me semblerait plus pertinent de modifier l'intitulé de cet article afin de faire preuve d'honnêteté et de transparence vis-à-vis de nos concitoyens. La vérité est que cet article 3 est un véritable tapis rouge pour les employeurs, afin, une nouvelle fois, de leur permettre de payer moins d'indemnités en cas de licenciement abusif.

Le taux de chômage extrêmement important de notre pays serait dû en partie, selon vous, à ces indemnités trop élevées ? Mais qui peut croire à cette argumentation ? Nous entendons toujours la même rengaine : « Il faut baisser le coût du travail pour libérer le travail », et ce, toujours, au détriment des mêmes, de la protection des salariés. Vous refusez de voir que le travail est avant tout source de richesse et que le problème est plutôt le coût du capital. Cela fait des décennies que les gouvernements successifs mettent en place

au moment de la rupture du contrat de travail. Toutes les mesures prévues sont autant de régressions : plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduction des sanctions prononcées contre l'employeur en cas d'irrégularité dans la procédure de licenciement, diminution des délais de recours contentieux pour les salariés, réduction du périmètre d'appréciation des difficultés économiques, allégement de l'obligation de reclassement. Parallèlement, l'article 3 prévoit d'accroître la flexibilité des contrats de travail, en élargissant les possibilités de recourir au CDI de chantier et en dérégulant les contrats courts, CDD, intérim. Pour toutes ces raisons, je propose de supprimer cet article.

habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances un certain nombre de mesures en faveur desquelles le Sénat s'est déjà prononcé à plusieurs occasions au cours des dernières années.

à un encadrement des dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une révision du périmètre d'appréciation de la cause économique d'un licenciement. Les amendements suivants nous donneront l'occasion de revenir en détail sur les différents éléments de l'article 3,

partisan du libéralisme ... L'article 3 aborde largement l'épineuse question des licenciements économiques. Mme la ministre nous assure qu'elle compte en revoir les modalités, notamment la question du périmètre d'appréciation des difficultés La commission des affaires sociales a réécrit cet article d'une façon qui me convient. J'espère qu'un compromis sera trouvé, car il faut à tout prix simplifier les règles. Le juge ne doit pas être en capacité d'apprécier la décision de mettre en oeuvre des licenciements économiques autrement qu'au travers de cette question du périmètre.

qui évoluent beaucoup plus rapidement que notre droit, de manière à favoriser les embauches. Toutes ces mesures vont dans le sens d'une plus grande flexibilité. Je répète que cette souplesse permettra des embauches, car les entreprises sauront que le droit du travail leur permet de s'adapter aux réalités de leur marché.

S'ils avaient créé des entreprises, risqué leurs biens pour les faire naître, pour les faire vivre, ils ne considéreraient pas que la multiplicité des règles, des instances, des représentants et des procédures est une sécurité pour les salariés.

du salarié. Je trouve que ce n'est pas du tout précariser les salariés ; c'est tout à fait les respecter ! Je ne vois pas où est le problème.

pour motif économique ou toute suppression d'emplois sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l'entreprise a constitué des réserves ou réalisé un résultat net ou un résultat d'exploitation positif au cours des deux derniers exercices comptables. « Est également dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d'emploi sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l'entreprise a, au cours des deux derniers exercices comptables, distribué des dividendes ou des stock-options ou des actions gratuites ou procédé à une opération de rachat d'actions. » Vous l'aurez compris, mes chers collègues, cet amendement vise à interdire les licenciements économiques dits « boursiers », dont l'unique objectif est l'augmentation de la rentabilité financière de l'entreprise. Cet amendement

Depuis la loi dite « El Khomri », une entreprise peut enclencher des licenciements économiques dès lors que ses commandes ou son chiffre d'affaires affichent une baisse. Seule exigence, un

ministre, va donc plus loin. Vous proposez, par exemple, de rendre négociable, au niveau de l'entreprise, et donc en amont, la motivation économique des licenciements.

Le code du travail doit être un outil de préservation de l'emploi et non d'amplification du chômage. Enfin, et c'est crucial, nous proposons de graver dans le marbre de la loi la jurisprudence

Nous y trouvons l'élément matériel- suppression ou transformation d'emplois ou modification du contrat de travail -, le périmètre d'appréciation, l'élément causal et ses quatre critères- difficultés économiques, mutation technologique, réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et cessation d'activité. La jurisprudence est bien établie sur ce sujet.

Vous proposez aussi de préciser que le licenciement doit être décidé en dernier recours par l'employeur. Toutefois, celui-ci est déjà soumis à une obligation préalable de recherche de reclassement et doit formuler des offres écrites précises individuelles aux salariés.

Il s'agit de faire référence à l'article L. 2211-1 du code du travail qui dispose que les dispositions relatives à la négociation collective s'appliquent aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés, aux établissements publics à caractère industriel et commercial, aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Par coordination avec sa position sur l'amendement n° 198, la commission émet un avis de sagesse positive

La connaissance du droit est un marqueur fort dans notre pays entre ceux qui ont le temps et les compétences pour développer une expertise juridique ou les moyens de s'attacher cette expertise, et les autres, laissés pour compte dans leur ignorance, stigmatisés et isolés. L'alinéa 3 de l'article 3 dont nous discutons constitue une avancée en ce qu'il charge l'autorité administrative de faciliter l'accès à l'ensemble des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles opposables à un salarié et à son profit, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut se prévaloir des informations obtenues dans ce cadre.

peuvent être d'une grande complexité. Il est indispensable que l'explication soit assurée de la façon la plus compréhensible possible, afin que chaque travailleur puisse pleinement prendre connaissance de tous les éléments, quel que soit son niveau de compétence juridique ou cognitive. Le niveau de compréhension juridique d'une personne n'est pas le seul frein à la compréhension du droit. Il convient de prendre en compte l'ensemble des situations de handicap de communication, que ce soit l'illettrisme, les troubles neurodéveloppementaux ou les déficiences intellectuelles, souvent non visibles. Pour pallier ces difficultés assez fréquentes, mon amendement tend à suggérer l'utilisation du français facile à lire et à comprendre, le FALC. Il s'agit d'une méthode reconnue, garantissant la bonne compréhension de l'information à délivrer,

l'intention des auteurs de cet amendement. Les sites publics d'information sur le droit du travail doivent être utiles et compréhensibles par l'ensemble des salariés et des employeurs. Comme le souligne Jean-Denis Combrexelle, le droit du travail est un droit complexe, réservé aux spécialistes, et, en même temps, un droit de proximité qui concerne des millions de nos concitoyens. Il faut en effet expliquer simplement des notions complexes, voire distinguer les niveaux d'explication sur le site. Le site offre offre un bon exemple de présentation pédagogique, avec des renvois vers des sites plus détaillés. Je rappelle toutefois que les informations fournies par le site public et prévues à l'alinéa 3 pourront ensuite être opposables par le salarié ou l'employeur en cas de différend administratif ou juridictionnel. Il est donc capital que les informations soient précises.

le CIH, le comité interministériel du handicap, du 2 décembre 2016 a proposé que l'ensemble des exposés des motifs des projets de loi soit aussi

la continuité du précédent, qui a pour objet de s'assurer que l'ensemble de nos concitoyens puissent comprendre les informations mises à leur disposition concernant le droit applicable à leur situation professionnelle. professionnelle. Il vise à garantir l'accessibilité de ces informations au plus grand nombre. Si la mise à disposition de ces informations par voie numérique est aujourd'hui la meilleure garantie d'assurer cette accessibilité au plus grand nombre, il est toutefois nécessaire de construire cette plateforme en tenant compte de toute forme de handicap éventuel des futurs utilisateurs Lors de l'examen du projet de loi pour une République numérique au Sénat, nous avions déjà débattu de la mise en accessibilité des sites internet pour les utilisateurs malvoyants ou malentendants.

pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui oblige les sites en ligne de l'administration à être accessibles aux personnes handicapées. Cet article dispose en effet : « Les services de communication au public en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées. » Cette accessibilité concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique. Les recommandations internationales pour l'accessibilité d'internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne. Un décret du 14 mai 2009 a d'ailleurs été pris en ce sens pour créer un référentiel d'accessibilité des services de communication publique en ligne. Ma chère collègue, votre amendement est

l'accès des personnes en situation de handicap à la culture, en particulier à la pratique culturelle, n'est pas aujourd'hui pleinement assuré. Les mesures se sont concentrées sur l'accessibilité et le droit à la compensation.

La parole est à M. Maurice Antiste. Cet amendement de repli tend à supprimer les dispositions plafonnant les indemnités prud'homales à la charge de l'employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Introduite prétendument au nom de la « sécurisation des relations de travail », cette disposition accroît en réalité l'insécurité des travailleurs en facilitant les licenciements abusifs, l'employeur connaissant à l'avance le prix maximal de son manquement. Les facilités supplémentaires accordées aux employeurs dans la procédure que les nouvelles contraintes de délai imposées aux salariés vont dans le même sens. Pour ces raisons, nous demandons la suppression des alinéas 4 à 6

de cette réparation. C'est dire au juge : « Vous n'avez pas la capacité d'apprécier la situation ; vous devez vous en tenir à ce que vous dit la loi. » Cela n'est absolument pas acceptable ! Par conséquent,

En réalité, comme je le disais, vous permettez à l'employeur de licencier abusivement alors que vous condamnez le salarié ou la salariée à la règle de l'arbitraire. Comment un salarié réclamerait-il le paiement de ses heures supplémentaires ou remettrait-il en cause une directive susceptible de porter à sa santé ou même au bon fonctionnement de l'entreprise si, du jour au lendemain, il peut être mis à la porte sans cause réelle et sérieuse, sans pouvoir se défendre et sans avoir la possibilité de voir reconnu son droit à l'indemnisation

le Gouvernement introduit dans le présent projet de loi le plafonnement des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sorti par la porte lors de l'examen de la loi El Khomri- il était devenu indicatif à l'issue du processus législatif et politique -, le plafonnement des indemnités prud'homales revient aujourd'hui par la fenêtre. On constate la détermination du Président de la République sur ce sujet : les premières dispositions en la matière avaient été instaurées par la loi Macron, comme l'a dit Mme Bricq, et celui qui était alors ministre de l'économie n'était pas étranger à la première mouture de la loi El Khomri.

D'une part, elle s'oppose au principe de la réparation intégrale du préjudice- cela a été dit par M. Tourenne. Selon ce principe du droit privé, tout le dommage causé, mais rien que le dommage causé, doit être réparé. Par définition, il y a contradiction avec l'idée d'un plafonnement des indemnités.

c'est bien du licenciement abusif dont nous parlons -, sauf, bien entendu, dans les cas de harcèlement et de discrimination. Lors de la discussion générale, madame la ministre, vous avez déclaré : « Les dommages et intérêts vont d'un à quatre pour le même préjudice, selon la juridiction, d'où un sentiment d'iniquité. Entreprises comme salariés ont besoin de repères. » Je peux l'entendre ; pour autant, dans les faits, nous savons très bien que le juge prud'homal est relativement raisonnable. Par ailleurs, si l'objectif est d'éviter des disparités et de donner aux entreprises plus de visibilité, je pense que le barème indicatif mis en place par la loi El Khomri, lequel varie en fonction de l'âge, de l'ancienneté

ce qui compte, c'est la réparation intégrale. C'est bien là le principe qui doit dominer tout le reste ! Qu'un barème indicatif existe, pourquoi pas ? Mais le salarié a droit, lorsqu'il est injustement licencié, à une réparation intégrale

Il incombe à la représentation nationale d'être plus précise sur ce point important et de fixer un plafond de dommages et intérêts, sauf à donner au Gouvernement et aux partenaires sociaux un chèque en blanc. Il est en l'occurrence proposé d'inscrire un plafond de dix-huit mois de salaire dans la loi.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait mentionné expressément les situations de discrimination et de harcèlement. À la réflexion, limiter l'exclusion du référentiel à ces deux seuls cas nous semble un peu trop restrictif. D'autres situations correspondent aussi à des atteintes à des principes d'ordre public ou à des libertés fondamentales, sans pour autant se rattacher directement à des actes de harcèlement ou de discrimination. Ces situations doivent également pouvoir être exclues du barème : par exemple, le licenciement d'une femme enceinte, d'un représentant du personnel,

Existent aujourd'hui un barème facultatif devant le bureau de conciliation et un barème facultatif devant le bureau de jugement. Ces deux barèmes ne sont d'ailleurs pas pris en compte dans la pratique. Si un barème obligatoire

le Gouvernement veut alléger les obligations de l'employeur en matière de motivation des licenciements et diminuer les sanctions en cas d'irrégularité de la procédure de licenciement. La commission des affaires sociales y a ajouté la reconnaissance, pour l'employeur, » : celui-ci serait autorisé à rectifier dans la lettre de licenciement les irrégularités de procédure et de motivation mineures qui sont sans incidence sur la cause réelle et sérieuse du licenciement. Ces mesures, qui transcrivent une demande récurrente des organisations patronales, remettraient en cause des protections fondamentales des salariés en autorisant une rectification de la part de l'employeur. La meilleure preuve de

que soient assouplies les exigences de motivation nécessaires et suffisantes applicables aux décisions de licenciement. Ainsi, l'absence de mention de la suppression du poste dans une lettre de licenciement économique

L'article 3 prévoit d'adapter les règles de procédure et de motivation applicables aux décisions de licenciement ainsi que les conséquences à tirer du manquement éventuel à celles-ci, en amont ou lors du recours contentieux. Il est clair, madame la ministre, que la motivation de la lettre de licenciement est un exercice jugé parfois difficile. Pour autant, il est nécessaire que le salarié connaisse les motifs de son licenciement. C'est ce qui lui permet de préparer sa défense s'il considère que ce licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. La commission des affaires sociales a souhaité reconnaître à l'employeur une forme de droit à l'erreur : celui-ci pourrait notamment corriger des irrégularités mineures de motivation. l'étude d'impact annexée au projet de loi indique que sur une centaine de décisions récentes, l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement est un motif très souvent mis en avant par les salariés dans les griefs justifiant la procédure contentieuse. insuffisance est rarement retenue par les juridictions. Par ailleurs, d'après l'étude d'impact, il serait envisagé d'établir un modèle type de lettre de licenciement au moyen d'un formulaire CERFA qui permettrait de sécuriser l'employeur sur le plan formel, pour l'aider à énoncer avec suffisamment de précision le ou les motifs de sa décision de licenciement. Nous proposons donc de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

La première porte sur les conditions dans lesquelles le juge apprécie, en cas de pluralité des motifs, c'est-à-dire lorsque plusieurs motifs sont invoqués, la réalité de la cause réelle et sérieuse. Dans un arrêt du 3 février 2016, la Cour de cassation a déterminé à quelles conditions un motif pouvait à lui seul entraîner la nullité du licenciement.

de petites entreprises qui ont mal formulé les termes d'un CDD sans que le juge considère qu'un problème se pose sur le fond : il s'agit d'une erreur formelle. En effet, certaines irrégularités de procédure en matière de conclusion des contrats à durée déterminée,

Comme vous l'avez rappelé à l'Assemblée nationale, madame la ministre, il est difficile d'expliquer au salarié ou à la petite entreprise que le délai de recours est d'un an pour les licenciements économiques collectifs et de deux ans pour les licenciements économiques individuels. Il nous faut rendre le droit plus lisible et plus accessible. C'est pourquoi le projet de loi prévoit d'harmoniser les délais de recours contentieux concernant la rupture du contrat de travail, afin de clarifier le régime juridique applicable. C'est là une très bonne chose, bien que ce sujet s'avère particulièrement sensible dans le cadre des concertations menées avec les partenaires sociaux. Si une harmonisation nous semble souhaitable, nous ne saurions, en revanche, soutenir la proposition de la commission des affaires sociales, qui suggère de réduire au moins de moitié le délai de recours en cas de licenciement économique,

Morhet-Richaud. La baisse des délais de prescription doit être envisagée globalement dans un souci de sécurité juridique. Il serait ainsi judicieux de prévoir un délai de prescription de deux ans, au lieu de trois, en matière de salaire. L'amendement n° 170 La prescription a pour objet de sécuriser les relations juridiques. Cette diminution de la prescription doit être envisagée pour tous les licenciements et non uniquement pour les licenciements économiques.

à supprimer le référentiel obligatoire pour fixer l'indemnité sans cause réelle et sérieuse. À notre sens, ce référentiel est très attendu par les employeurs. Cet amendement vise en outre à supprimer le droit à l'erreur des employeurs lors des procédures de licenciement

ce qui crée de l'incertitude, aggravée par la grande disparité des pratiques des juges sur le territoire. Le Conseil constitutionnel a accepté le principe du barème. Dans sa décision du 5 août 2015, il a en effet considéré que le principe même d'un encadrement de l'indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse n'était pas contraire à la Constitution : en cherchant à « assurer

Je rappelle que le juge restera toujours libre d'individualiser l'indemnité en respectant le plafond fixé. Il pourra ainsi retenir, par exemple, le quart, la moitié ou les trois quarts du plafond, selon le préjudice subi. Je rappelle aussi que les cas de harcèlement

ont adopté un encadrement de l'indemnité, comme le rappelle l'étude de législation comparée du Sénat annexée au rapport de la commission. Ainsi, en Belgique, le plafond de l'indemnité est compris entre trois et dix-sept semaines de rémunération.

L'amendement n° 119 vise, selon la commission des affaires sociales, à autoriser le juge à verser à un salarié des dommages et intérêts indépendamment du barème obligatoire s'il remplit certains critères. Il revient donc à réduire la portée et l'ambition du référentiel, qui est de verser une seule et unique indemnité pour les dommages et intérêts liés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si l'on multiplie les indemnités parallèles, le référentiel perd de son intérêt. J'ajoute que le référentiel devrait au moins comporter un critère, celui de l'ancienneté du salarié. Mais le Gouvernement pourra en rajouter d'autres dans l'ordonnance s'il le souhaite. Enfin, les critères mentionnés dans l'amendement seront, bien entendu, utilisés par le juge pour individualiser l'indemnité, sans dépasser le plafond fixé dans le référentiel. La commission émet donc un avis défavorable

économiques, la loi Macron, qui instituait un référentiel obligatoire pour fixer l'indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais qui a été censuré par le Conseil constitutionnel, prévoyait un cumul avec les indemnités de licenciement.

son plafond est fixé à vingt et un mois et demi pour un salarié ayant plus de quarante-trois ans d'ancienneté. Un référentiel indicatif en phase de conciliation quant à lui, un plafond de vingt-quatre mois pour les salariés ayant plus de trente ans d'ancienneté. Un référentiel impératif en phase de jugement, qui figurait à l'article 266 de la loi Macron avant sa censure par le Conseil constitutionnel, prévoyait même un plafond de pour les salariés ayant plus de dix ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 300 salariés. L'étude de législation comparée du Sénat, qui a été annexée au rapport de la commission, montre que des plafonnements sont fréquents en Europe. comme vous avez annoncé votre souhait de relever les indemnités légales de licenciement, qui sont parmi les plus faibles d'Europe, on pourrait peut-être accepter de baisser un peu le plafond maximal du référentiel obligatoire.

n° 228, le Gouvernement souhaite que le référentiel ne s'applique pas si le licenciement est entaché par une faute de l'employeur d'une particulière gravité. Ce faisant, il souhaite augmenter le nombre des cas dans lesquels le référentiel ne s'appliquera pas. Le texte prévoit actuellement seulement deux exceptions : la discrimination et le harcèlement. Mais l'ordonnance pourra en prévoir d'autres. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. » L'habilitation demandée par le Gouvernement ne remettra pas en cause ce principe. Elle autorisera seulement l'employeur à rectifier des erreurs de procédure secondaires, notamment sous le contrôle du juge, à condition que l'employeur puisse effectivement s'appuyer sur une cause réelle et sérieuse de licenciement. J'attire votre attention sur le fait que le législateur a déjà reconnu l'an dernier une forme de droit à l'erreur à l'administration en matière de plan de sauvegarde En effet, en cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative est autorisée à prendre une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de quinze jours.

effet de supprimer l'apport de la commission à l'alinéa 4, qui visait à encadrer la concertation des partenaires sociaux, dans le prolongement des pistes évoquées dans l'étude d'impact. Mais, dans le même temps, il est proposé d'élargir l'habilitation à deux sujets importants. Le premier concerne les motifs contaminants dans une procédure de licenciement. Le professeur Jean-Emmanuel Ray, que nous avons auditionné, a souligné que la jurisprudence de la Cour de cassation pouvait avoir de graves conséquences sur les employeurs.

qui fait tomber toute une procédure de licenciement, même si elle repose sur une cause réelle et sérieuse par ailleurs. Le second élargissement consiste à mieux encadrer les cas autorisant une requalification d'un CDD en CDI. Pour toutes ces raisons,

de l'alinéa 6, relatif à la réduction des délais de recours en cas de licenciement. Les auteurs de cet amendement rappellent avec raison la très forte hétérogénéité des délais pour contester un licenciement, de deux mois à cinq ans. Mme la ministre y a fait référence tout à l'heure. Une

du délai de contestation d'un licenciement économique. Un tel délai paraît suffisant pour un salarié pour savoir s'il veut former un recours. Augmenter les délais de prescription n'apporte pas toujours de protection supplémentaire aux salariés. En revanche, cela aboutit systématiquement à créer de l'incertitude pour les employeurs et à nuire à l'attractivité de notre territoire. La commission émet donc un avis défavorable

proposent d'aller plus loin que le texte de la commission. Si je partage l'objectif de réduction et d'harmonisation des délais de contestation, je souhaite que nous nous en tenions à la rédaction de la commission, en espérant que le Gouvernement et les partenaires sociaux trouvent un terrain d'entente pour réduire et